monsieur le président.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

de la commission chargée de la certification professionnelle ne crée pas de difficulté supplémentaire en soi dans la procédure d'enregistrement des certifications, il importe néanmoins d'assortir ce dispositif de conditions de transparence et de sincérité à l'égard des organismes certificateurs. L'amendement n° 372 vise donc à ce que l'avis conforme rendu par cette commission de France compétences s'établisse sur des critères objectifs et transparents. L'avis conforme- ou son refus -doit également être motivé et notifié à l'organisme certificateur requérant. Par l'amendement n° 373, nous prévoyons un dispositif miroir en matière de transparence pour les certifications professionnelles. Les amendements

et de différenciation, ce qui concourt à une perte de visibilité et de qualité des formations ? Concernant l'amendement n° 515 rectifié, l'article 14 prévoit de remplacer la Commission nationale de la certification professionnelle par une commission chargée de la certification professionnelle au sein de France compétences. Intégrer cette commission au sein de France compétences permettra d'assurer une cohérence entre la certification et les besoins en compétences que France compétences aura identifiés. La commission des affaires sociales a renforcé la gouvernance quadripartite de France compétences afin qu'elle ne soit pas seulement une agence de l'État. Par ailleurs, un décret précisera la composition et les attributions de cette nouvelle commission afin qu'elle conserve son indépendance. Je considère que cet amendement est satisfait à

L'amendement rédactionnel n° 40 rectifié tire les conséquences du changement de statut juridique de France compétences opéré par l'Assemblée nationale : avis favorable. Merci Les amendements n 372 et 373 n'apportent pas, selon nous, une telle plus-value au dispositif qu'ils mériteraient de compléter la loi. Un décret est prévu pour déterminer les modalités d'enregistrement des diplômes, titres et certificats.

des amendements identiques n 19 rectifié et 105 rectifié, si l'article 14 pose le principe d'une coconstruction des certifications professionnelles en associant les branches professionnelles, il est important de maintenir une régulation de la certification professionnelle. Par conséquent, France compétences pourra demander que des correspondances soient mises en place entre les certifications et en retirer certaines des répertoires de la certification professionnelle, afin de s'assurer de l'homogénéité et de la cohérence des certifications entre elles. Je demande donc le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.

L'accord national interprofessionnel du 22 février prévoit que les partenaires sociaux ont la responsabilité des référentiels métiers. Les branches assurent par ailleurs, au niveau professionnel et interprofessionnel, le pilotage des certifications de branche et interbranches. Or le projet de loi ne précise pas le rôle des branches professionnelles. Il convient donc de rappeler que les référentiels d'activité et de compétences sont élaborés par les branches. L'amendement n° 693 rectifié,

visent à compléter des dispositions générales pour l'ensemble des certifications professionnelles qui prévoient que toutes les certifications professionnelles seront définies par des référentiels. Pour les diplômes et les titres, ces référentiels seront élaborés par les commissions professionnelles consultatives, ou CPC. Les certificats de qualification professionnelle seront, quant à eux, élaborés par les branches.

Cet amendement, dans un souci de souplesse et d'adaptation, tend à ce que les référentiels de diplômes et titres à finalité professionnelle puissent être adaptés aux caractéristiques et spécificités de chaque territoire régional. L'amendement n° 612, chapitre entend refondre le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels, notamment par un travail concerté avec les partenaires sociaux. L'esprit du projet de loi suppose ainsi une coconstruction en étroite relation avec les entreprises locales. Aussi, dans un souci de souplesse et d'adaptation, nous proposons, par le présent amendement, que les référentiels de diplômes et titres à finalité professionnelle puissent être adaptés aux réalités du terrain par la prise en compte des caractéristiques et spécificités de chaque territoire. ? Nous entrons là dans une délicate problématique ... Nous ne percevons pas la nécessité d'adapter ces référentiels aux spécificités des territoires.

notamment en conditionnant le financement du compte personnel de formation à l'enregistrement au RNCP ou au répertoire spécifique. Dans le cadre de la démarche qualité que nous souhaitons promouvoir, le caractère systématique de cette demande

L'exercice de cette profession ne bénéficie cependant d'aucune base légale permettant de garantir le haut niveau de qualité des prestations des architectes d'intérieur et d'apporter la reconnaissance de diplômes sanctionnant cinq années d'études. Aux termes d'un travail de concertation mené avec les pouvoirs publics en 1996, les architectes d'intérieur exercent leur activité conformément à la « charte relative à la formation des architectes d'intérieur » élaborée par la direction de l'architecture du ministère de la culture.

L'aboutissement de ce travail, attendu dans les prochaines semaines, consacrera conjointement le haut niveau des formations dispensées et le travail de qualité des professionnels. Il est à noter que la reconnaissance de l'activité des architectes d'intérieur est un engagement gouvernemental pris il y a deux ans devant la Haute Assemblée. La reconnaissance du titre d'architecte d'intérieur nécessite l'adoption d'une disposition législative. On signalera que la création de ce titre d'architecte d'intérieur ne pose pas de difficulté aux architectes et au Conseil national de l'ordre des architectes, qui soutient cette création. Au contraire, les architectes désireux d'exercer leur art sous le titre d'architecte d'intérieur pourront le faire sans condition de réciprocité, car il convient naturellement de continuer à assurer la plus grande protection du titre d'architecte.

la commission ? Cet amendement vise à créer une disposition spécifique pour les architectes d'intérieur qui revient à réglementer l'accès à cette profession, sans que cela nous paraisse justifié.

seulement 35 % d'entre elles sont en situation d'emploi. Pour favoriser leur insertion professionnelle, la circulaire autorise les recteurs à délivrer aux jeunes en situation de handicap une attestation de compétences quand ces derniers ne sont pas en capacité de valider la qualification à laquelle ils aspiraient. Clairement, cette circulaire partait d'une bonne intention et l'adoption d'un amendement à ce texte tendant à la généraliser répondait à la même problématique.

Elle pourrait même constituer un affaiblissement de l'ensemble du système de qualification. Plutôt que d'abaisser le niveau de formation des personnes en situation de handicap, il nous semble essentiel de réunir l'ensemble des conditions pour qu'elles puissent atteindre la qualification. Cela doit permettre une meilleure insertion, mais aussi favoriser la poursuite d'études, car si le nombre d'étudiants handicapés a triplé en dix ans, ils ne sont que 23 000, alors que l'on compte 350 000 scolaires en situation de handicap. Concrètement, cela implique qu'une part importante des enfants en situation de handicap n'arriveront pas à atteindre l'enseignement supérieur, alors même que la massification de ce niveau d'études est un enjeu sociétal au vu des défis techniques et technologiques

qu'une solution d'urgence, et non une solution viable à long terme. C'est pourquoi nous proposons de réunir les conditions de la réussite des élèves en situation de handicap en complétant le projet personnel de scolarisation

des affaires sociales de modifier l'article 14 afin que les personnes handicapées ayant suivi une formation puissent recevoir les blocs de compétences qu'elles ont validés si elles ne peuvent pas obtenir le diplôme ou le titre visé. amendement supprime cette possibilité. Il se limite à préciser que le projet personnalisé de scolarisation devra prendre en compte le passage des examens, ce qui est déjà couvert par la possibilité d'aménagement des modalités de déroulement de la scolarité.

Faire négocier les organisations syndicales participe de la sensibilisation des entreprises et d'un accompagnement des TPE-PME, qui représentent 99,8 % des entreprises en France. Ces négociations permettront d'aborder l'ensemble du parcours de vie des proches aidants dans l'entreprise. Les branches pourraient notamment décider de leur donner une priorité d'accès à une formation professionnelle au retour d'une longue absence ou de faciliter le recours au télétravail. télétravail. Notre ancienne collègue Dominique Gillot a récemment souligné, dans un rapport remis à Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, qu'une réflexion devrait être menée dans ce sens. Il nous appartient de créer les conditions d'une meilleure articulation entre vie professionnelle et exercice de la solidarité pour tous les salariés, quelle que soit l'entreprise, afin que celui-ci ne soit plus synonyme de renoncement et d'inégalité professionnelle.

L'amendement visait à l'origine à rendre obligatoire, au niveau des branches et des entreprises, la négociation sur la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des proches aidants.

manière générale, la commission ne souhaite pas modifier les règles de la négociation collective, qui ont été refondues par la loi Travail du 8 août 2016 et par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017,

Corinne Féret, sur l'article. L'article 15 traite notamment de la nouvelle répartition des rôles entre acteurs de l'apprentissage et de la formation professionnelle.

En effet, pilotes de l'apprentissage et de la formation professionnelle, les régions se voient retirer la compétence en matière d'apprentissage. Leurs moyens seront très limités, alors même qu'elles assument, avec les partenaires sociaux, des responsabilités centrales en termes de développement économique, de formation et d'orientation.

dont l'implantation pourrait ne répondre qu'aux seules contingences économiques, et le développement d'une vision « adéquationniste » de la formation, avec une possible baisse de sa qualité, car on peut on peut s'interroger sur la capacité des branches à appréhender seules les enjeux à l'échelle de l'ensemble des territoires. Seules les branches les mieux organisées auront les moyens financiers et humains de le faire.

Ces centres disposent d'un accès à une base de données nationale regroupant des informations sur les différentes formations. Transmettre cette compétence aux régions, c'est leur laisser la possibilité d'effectuer des arbitrages financiers en fonction de leurs priorités, ce qui est je le rappelle, n'est pas envisagée de la même façon par toutes les régions et n'est pas toujours leur priorité. Or tous les élèves et tous les étudiants devraient pouvoir avoir accès aux mêmes informations en matière de formation et recevoir des conseils d'égale qualité,

pas le centralisme démocratique,

Présenté comme devant renforcer les liens avec le monde de l'entreprise, le transfert de l'apprentissage aux branches professionnelles, et donc le dessaisissement des régions, ne pourra que nuire à cette filière dont le développement est essentiel pour l'accès de nos jeunes à l'emploi. les premières lois de décentralisation, les régions se sont vu confier la compétence en matière de formation professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi, ainsi que les politiques d'apprentissage. Les lois successives ont renforcé leurs pouvoirs dans ces domaines. Le Gouvernement, en écartant les régions, nie le rôle qu'elles ont joué et jouent de plus en plus dans le développement de l'apprentissage. Les branches professionnelles, qui sont appelées à reprendre la quasi-totalité de leurs missions, sont loin d'être présentes sur tous les territoires, certaines n'ont même aucune culture de l'apprentissage, d'autres sont en cours de restructuration. De plus, la compétence de régulation par la péréquation territoriale dont héritent les régions ne mobilisera pas assez de moyens pour leur permettre d'intervenir efficacement.

Aussi le présent amendement vise-t-il à rétablir la compétence générale des régions en matière d'apprentissage. Cet amendement n'est pas compatible avec les autres dispositions du texte concernant l'apprentissage. En effet, l'article 11 prévoit que les CFA seront créés sans l'aval des régions. L'article 19 prévoit le financement de l'apprentissage au contrat par les opérateurs de compétences selon un niveau de prise en charge fixé par les branches professionnelles. Par conséquent, la région ne pourra plus, dans ce nouveau schéma, définir et mettre en oeuvre seule la politique de l'apprentissage et adopter la carte régionale des formations professionnelles initiales. C'est pourquoi, madame la ministre, dans ce nouveau schéma, la commission a toutefois renforcé le rôle des régions, qui pourront élaborer une stratégie des formations en alternance et conclure des conventions d'objectifs et de moyens avec les CFA qu'elles soutiendront financièrement.

les régions pour donner davantage de compétences aux branches. Vous avez trouvé un accord avec une partie du MEDEF, avec quelques branches qui sont certainement en

dans un pays unitaire- la France n'est pas une fédération -, le fait que des compétences soient décentralisées en vue de la réalisation d'un certain nombre de missions de service public ne prive pas l'État

avec la région comme organisateur. Vous le savez tous et toutes : une loi va arriver, qui confiera le pilotage non plus aux régions, mais aux entreprises et aux branches professionnelles. [ ...] D'habitude, un élu, quand on lui enlève ses compétences, est le premier à râler Pourquoi je ne râle pas ? Parce que je pense que le nouveau système peut être plus efficace. Je pense que le nouveau système, en partant du besoin des entreprises et en confiant la responsabilité aux entreprises, peut nous permettre d'avoir plus de jeunes en apprentissage, donc moins de jeunes au chômage, et des entreprises ayant plus

Contrairement aux engagements pris par le Premier ministre le 9 février dernier, la mise en place d'un schéma rassemblant les conventions d'objectifs et de moyens signées avec les branches professionnelles et donnant une perspective pluriannuelle au développement de l'alternance, notamment en matière d'investissements, en fonction des perspectives économiques des territoires et du projet économique régional ne figure pas dans le projet de loi. L'ensemble du débat sur l'apprentissage montre que donner les clefs soit aux régions, soit aux branches n'est pas totalement satisfaisant. Sans remettre en cause le principe de libre ouverture des CFA et des sections d'apprentissage, les auteurs de cet amendement proposent de définir les prémices d'une compétence partagée des régions et des branches en matière d'apprentissage. Il s'agit de mutualiser les points forts des acteurs pour atteindre l'objectif de souplesse et de réactivité fixé par le Gouvernement.

de répartir les investissements selon une logique d'aménagement du territoire, d'organiser la complémentarité des lycées professionnels et des CFA, plutôt que leur mise en concurrence déloyale, et de promouvoir cette logique dans la perspective d'un développement des campus des métiers et des qualifications.

et de développer les campus des métiers et des qualifications.

Cette stratégie permettra à chaque région d'identifier les besoins en matière d'offre de formation professionnelle initiale sur son territoire et de définir sa politique de soutien à l'apprentissage en conséquence.

Il y a donc lieu de s'orienter vers une unification et une rationalisation de la commande de formations. À cette fin, le présent amendement vise à instaurer une compétence de principe de la région pour l'ensemble des formations individuelles et collectives, tout en maintenant la possibilité d'une intervention de Pôle emploi dans le cadre d'une convention conclue avec la région.

Il peut être utile d'unifier les règles d'achat de formations, qu'elles soient individuelles ou collectives, et d'associer les régions dans tous les cas. Toutefois, la rédaction de l'amendement n°

M. Daniel Chasseing. Cet amendement rappelle le rôle important des branches dans l'information sur les besoins des entreprises. L'accord interprofessionnel du 22 février dernier a consacré le rôle des branches professionnelles dans l'expression des besoins des entreprises l'information sur les métiers. À ce titre, les commissions paritaires de branche, telles que les commissions paritaires nationales et régionales de l'emploi, ont pour mission de définir les axes prioritaires en matière de formation professionnelle, d'alternance et de certifications professionnelles de la branche, correspondant aux besoins en emplois et compétences, et d'orienter les moyens mis en oeuvre pour leur développement. Nous proposons de reprendre cette précision, afin d'assurer un pilotage de l'emploi et de la formation professionnelle à tous les niveaux. Quel est l'avis de la La commission estime qu'il ne faut pas trop bouleverser le paysage conventionnel avant qu'il ne parvienne à se restructurer. En outre, le projet de loi confie déjà aux branches professionnelles un rôle important en matière d'apprentissage et pour la définition des diplômes et des titres ; elles pourront identifier les besoins en compétences des entreprises. C'est pourquoi nous émettons un avis défavorable sur l'amendement. même avis que la commission

les moyens mobilisés au titre du droit commun restent quantitativement et qualitativement insuffisants compte tenu des enjeux et le recours aux moyens spécifiques, mal ciblé. [ ...] La priorité que devrait constituer l'accès dans des conditions de droit commun au milieu ordinaire de travail est insuffisamment prise en compte. » Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement

dans un marché concurrentiel. Or aucun critère d'intervention des régions n'est défini. La justification d'aménagement du territoire ou de développement économique reste confuse. Le renvoi à l'article L. 6332-14 du code du travail permet uniquement de fixer les critères qui doivent être pris en compte par les opérateurs de compétences pour l'élaboration du niveau de prise en charge. Le cadre juridique n'est donc absolument pas sécurisé pour les régions, notamment au regard du droit européen sur l'intervention de la puissance publique

de modifier la rédaction du 1° de l'article L. 6211-3 du code du travail pour permettre une autre utilisation des dépenses de fonctionnement des régions et élargir le champ d'action et d'intervention la possibilité d'abonder les dispositifs d'aide aux apprentis et de mettre en oeuvre des actions de valorisation de l'apprentissage dans un cadre juridique sécurisé, sans risque au regard du droit européen. L'adoption de cet amendement permettrait de cibler des dépenses qui relèveront encore du champ des compétences régionales.

il paraît opportun, dans la mesure où les régions sont des collectivités territoriales et non des services déconcentrés de l'État, de prévoir que le montant de ces dépenses, tant en fonctionnement qu'en investissement, fera l'objet d'un débat annuel en conseil régional, sur le fondement d'un rapport présenté par l'exécutif et transmis pour

dont le rôle est réaffirmé par le projet de loi, reconnaît les besoins des branches professionnelles et la réalité des territoires. L'objectif de cet amendement est de permettre la prise en compte des territoires pour une mise en cohérence au regard des besoins des entreprises, en fonction des spécificités territoriales et de l'ancrage territorial des entreprises. Je sais bien que l'on ne fait pas une politique à coup d'exemples, et qu'à tout exemple on peut opposer des contre-exemples.

facilitent l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers non seulement dans les domaines de la transition écologique et énergétique, mais aussi dans celui du numérique, filière d'avenir par excellence.

Les opérateurs de compétences agiront pour le compte des branches adhérentes. Ces dépenses étant une faculté de la région au regard des besoins identifiés, il est important que les conventions d'objectifs et de moyens restent

de plan régional de développement des formations professionnelles, identifieront l'émergence de nouvelles filières économiques et de nouveaux métiers, il semble évident qu'elles le feront notamment dans le domaine du numérique,

et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes. Toutefois, se limiter à ce seul niveau contractuel apparaît insuffisant. Il convient en effet, eu égard à la capacité des régions de contribuer au financement des formations en alternance, que ces dernières puissent également conventionner

Le texte tel qu'amendé par la commission prévoit déjà que, au titre des dépenses régionales de soutien aux CFA, les régions pourront conclure des conventions d'objectifs et de moyens avec ces Toutefois, ces dépenses ne sont pas destinées à soutenir financièrement les lycées professionnels, qui dépendent du ministère de l'éducation nationale. Il n'y a donc pas lieu que les régions concluent de telles conventions avec ces lycées.

France compétences, qui disposera des fonds de péréquation, il importe que les régions puissent apprécier les besoins des CFA de leur territoire. À cette fin, il convient de prévoir que chaque année, avant le 30 juin, les CFA transmettent à la région leurs documents comptables et financiers.

des centres subventionnés. Par ailleurs, France compétences sera administrée par des représentants des régions et attribuera aux régions les fonds destinés à majorer la prise en charge par contrat d'apprentissage selon des critères définis à l'issue d'un dialogue avec les régions et fixés par décret.

est ainsi libellé : La parole est à M. Martin Lévrier. La commission des affaires sociales du Sénat a souhaité préciser que, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles, la région élaborera une stratégie régionale pluriannuelle des formations en alternance. Cette stratégie sera élaborée en lien avec les acteurs économiques et les partenaires sociaux des territoires. Le projet du Gouvernement est bien de confier davantage aux entreprises la gestion du système d'apprentissage afin de sortir du modèle issu de la loi de 2014, qui n'a pas fait ses preuves. ses preuves. Aussi convient-il de ne pas recréer un tel modèle en conditionnant l'initiative des branches professionnelles pour le développement de l'apprentissage au respect des obligations qui leur seraient fixées au travers des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles. Un tel système serait susceptible de les empêcher de se saisir pleinement de leur compétence en matière de développement de l'apprentissage, et donc de freiner ce développement. Quel Sans remettre en cause les prérogatives accordées aux branches professionnelles et aux opérateurs de compétences en matière d'apprentissage, la commission a tenu à ce que ces acteurs tiennent compte de la stratégie des formations en alternance qui sera élaborée par chaque région. La région ayant une connaissance des bassins d'emploi et des besoins de formation dans son territoire, elle conservera une capacité de financement s'agissant de l'apprentissage. Il est donc important qu'il y ait une prise en compte du rôle de chaque acteur pour le développement de l'apprentissage. L'avis est défavorable.

qui est de transformer en profondeur l'apprentissage pour responsabiliser chaque acteur au bon niveau d'intervention, en donnant la priorité aux entreprises et aux apprentis.

professionnelles, les CPRDFOP, qui existent déjà et permettent de définir une vision globale en matière d'orientation et de formation professionnelles incluant l'apprentissage, plutôt que de rajouter un schéma spécifique en matière d'apprentissage.

Comme indiqué précédemment, les CFA seront librement créés et établir une carte des formations en apprentissage ne sera donc plus possible.

par les régions en 2018 et en 2019 et visant à déterminer les coûts moyens des contrats d'apprenti pour assurer la transition avec le nouveau dispositif et permettre aux régions de maintenir un niveau suffisant d'investissement dans l'ensemble des CFA. ainsi proposé que le rapport soit rendu avant le 15 juillet, au lieu du 1 mai, pour tenir compte de la date limite de vote des comptes administratifs, fixée au 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré. Cet amendement vise à donner plus de temps aux régions pour établir leur rapport sur les dépenses en matière d'apprentissage, qui nécessitera d'agréger de nombreuses données. L'avis est favorable. Très bien ! Quel

Dans un tel contexte, le maintien de la compétence des régions à titre dérogatoire et transitoire permettrait d'assurer la pérennité des dispositifs de formation existants tout en préparant sereinement la mise en oeuvre de la loi à partir du 1 janvier 2023,

? Les amendements n°382 et 558 rectifié tendent à repousser l'entrée en vigueur de l'article 15 au 1 janvier 2023 dans certaines collectivités d'outre-mer.

Le scrutin est ouvert.

cette volonté de recentralisation, tout comme nous nous opposons à celle de privatiser une politique publique en confiant aux seules branches professionnelles la responsabilité de l'apprentissage. branches professionnelles la responsabilité de l'apprentissage. Notre pays compte des centaines de branches professionnelles, à l'organisation très disparate : certaines regroupent quelques dizaines de salariés, d'autres plusieurs centaines de milliers. Alors qu'elles ne couvrent ni tous les métiers ni tous les Français, comment ces branches pourraient-elles faire mieux que dix-huit régions ?

Nous tenons à ce que les régions conservent un rôle ; tel est le sens du texte de la commission. Les branches professionnelles en joueront aussi un, dans le cadre de la définition du coût au contrat d'apprentissage. Ces amendements posent donc le principe de prérogatives partagées.

a pour objet de permettre à la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, de gérer les appels à projets émis dans le cadre du volet national du plan d'investissement dans les compétences. En effet, la CDC a une grande expérience en matière d'appels à projets dans le domaine de la formation et de l'insertion professionnelle, et elle exerce des missions d'intérêt général pour le compte de l'État et des collectivités territoriales. En outre, elle contribue au développement économique des territoires. Le ministère du travail restera bien

? Cet amendement vise à sécuriser la gestion des actions mises en oeuvre au titre du plan d'investissement dans les compétences, en en confiant la gestion à la Caisse des dépôts et consignations, à l'instar de ce qui a été prévu pour le programme d'investissements d'avenir. L'avis de la commission est bien entendu